pourquoi pas ?

Nous avons amorti la dette sociale et nous supprimons la CRDS.

la CRDS constitue aujourd'hui l'impôt sur le revenu le plus large de notre droit positif. À l'examen des documents financiers de la CADES, il semble que cette nouvelle consolidation assure pour environ une année et demie encore l'existence de la caisse comme des contributions qui l'alimentent, la CRDS ayant été rejointe pour partie par la CSG. Le tout, aujourd'hui, permet de totaliser plus de 15 milliards d'euros de recettes fiscales. Fin 2017, ces dernières ont dégagé un intéressant excédent permettant l'amortissement d'une partie de la dette sociale, qui atteignait alors 120 milliards d'euros

rapporteur général. Cet amendement a pour objet de transférer prioritairement à la CADES les déficits des branches et du fonds dont la trajectoire de solde rend le remboursement de la dette plus aléatoire. Dans cette perspective, la branche maladie et le fonds de solidarité vieillesse, le FSV, doivent pouvoir transférer leur dette en priorité. La branche famille devrait pouvoir financer ses déficits par elle-même. Quant à la branche vieillesse, elle n'a pas besoin de transférer de dettes à la CADES.

à cette caisse de financer la dette qui lui sera transférée en application de l'article 20. Enfin, il est expressément indiqué que la CADES percevra un produit supplémentaire de 5 milliards d'euros en 2023-

Il vise à abroger l'affiliation des élèves des lycées professionnels maritimes et des étudiants de l'École nationale supérieure maritime, l'ENSM, au régime des marins. Pour l'heure, ces élèves et étudiants ne relèvent pas du régime spécifique des étudiants,

Toutefois, le régime spécial des marins gère la caisse de retraite des marins du commerce, de la pêche et de la plaisance professionnelle. En adoptant cette disposition, on prive ce régime spécifique de nouveaux entrants. Je comprends la volonté que traduisent ces dispositions. Mais, dans cette période

Chasseing. Depuis l'an 2000, les médecins et les psychologues experts judiciaires sont qualifiés de collaborateurs occasionnels du service public, ou COSP, et

Cette situation affecte tout particulièrement les médecins légistes, les psychiatres et les psychologues, dont les honoraires au pénal sont tarifés. À l'heure où l'on constate une grave pénurie de médecins experts

amendement a pour objet de maintenir les experts relevant du régime général dans ce même régime quand ils sont requis, commis ou désignés par l'autorité judiciaire.

de sa population adhérente risque de déstabiliser durablement le régime complémentaire dont il s'agit et, plus largement, le régime de base des professions libérales ; au regard des effectifs, la CIPAV est la plus importante des sections professionnelles composant l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales. la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a prévu un mécanisme de compensation financière, lequel doit être organisé par une convention-cadre conclue entre les régimes concernés.

qui figurent à l'annexe 5. Ces « niches sociales », qui se sont multipliées depuis les années 1990, sont censées permettre d'atteindre des objectifs de politiques publiques,

aux grands patrons, que le Gouvernement chérit tant ... Or, vous le savez, ce projet de budget tout entier a été construit autour de l'idée de désendettement de la sécurité sociale. Lorsqu'on voit l'importance de ce manque à gagner pour notre sécurité sociale,

que ces exonérations sont de nature à favoriser la création d'emplois. Enfin, le comité de suivi du CICE lui-même a annoncé, dans son rapport de

Nous rejoignons tout à fait l'analyse du rapport de la commission des affaires sociales sur cet article : « Le rabotage dès à présent de la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale, dans des proportions très significatives et sans un quelconque accord du Parlement sur les principes devant régir, à l'avenir, les relations financières entre l'État et la sécurité sociale, est prématuré. C'est une manière édulcorée de pointer à nouveau ce que nous avons déjà affirmé dans les différentes travées de notre hémicycle : notre refus de la participation de la sécurité sociale à la prise en charge du renforcement des allégements généraux et du transfert des éventuels futurs excédents de la sécurité sociale vers les caisses de l'État. Deux problèmes majeurs sont devant nous : la situation critique de l'hôpital et la question de la perte d'autonomie. Si excédents il y a demain, ceux-ci devront être consacrés à ces enjeux d'avenir pour notre pays. la hausse de l'ONDAM, prévue pour les quatre années à venir à 2,3 %, permettra-t-elle de financer la réforme du système de santé présentée récemment par le Président de la République ? en cohérence avec la position que nous défendons depuis le début de ce débat, vise donc à supprimer cet article et, ainsi, à promouvoir l'autonomie financière de la sécurité sociale. La parole

décrit l'évolution de l'ONDAM pour les quatre années à venir. Pour l'année 2019, l'augmentation de l'ONDAM a été fixée à 2,5 %, soit une amélioration de 0,2 point par rapport à l'année 2018, ce dont le Gouvernement ne manque pas de se féliciter.

1,1 milliard d'euros sur le médicament, quasiment 2 milliards d'euros pour le régime général, à cause des faibles revalorisations des prestations sociales et des pensions de retraite- nous en avons beaucoup parlé hier -et presque 1 milliard d'euros pour les hôpitaux, dont tout le monde dit pourtant qu'ils se trouvent dans une situation extrêmement difficile.

L'avis du Gouvernement est évidemment défavorable. Nous nous opposons à la mesure et donc au réajustement du tableau, monsieur le rapporteur général.

de pompiers volontaires, créant une charge supplémentaire pour la sécurité sociale pouvant atteindre jusqu'à 500 millions d'euros à terme, selon notre compréhension de l'amendement adopté, dont plus de 100 millions d'euros pour l'année prochaine.

vous avez également choisi d'appliquer le barème de compétitivité renforcée au secteur du nautisme, aux services aéroportuaires, aux liaisons aériennes entre pays voisins, aux activités de comptabilité, de conseil aux entreprises, d'ingénierie et d'études techniques. Cela représente un coût d'au moins 200 millions d'euros. Vous avez, enfin, adopté un renforcement des exonérations des particuliers en outre-mer, pour un coût que nous ne savons pas déterminer. Vous avez souhaité étendre la mesure d'atténuation du franchissement des seuils de CSG, pour un montant de 100 millions d'euros

À cette facture, s'ajoutent 40 millions d'euros pour le renforcement des exonérations pour les chambres consulaires, 7 millions d'euros pour les porteurs de presse, 10 millions d'euros pour les médecins en cumul emploi-retraite et 10 millions d'euros pour l'abaissement à 8 % du taux de forfait social.

Monsieur le président, madame la ministre, ce ne sont pas mes amendements qui ont tant coûté, puisqu'aucun d'entre eux,

je vais mettre aux voix la troisième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. Je vous rappelle que, lorsque le Sénat n'adopte pas les dispositions de cette partie, la quatrième partie du projet de loi est considérée comme rejetée. Y a-t-il des demandes d'explication de vote ? ... Je mets aux voix l'ensemble je vais mettre aux voix la troisième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019.

Le scrutin est ouvert.

de qualité. À l'Assemblée nationale, le rapporteur général et vous-même avez précisé le dispositif : un développement des indicateurs après négociations en 2019, le recueil des indicateurs « à blanc puis leur intégration au modèle de financement la première année, financement dont la première année est fixée à 2020 pour les établissements de soins de suite et pour l'hospitalisation à domicile et à 2021 pour la psychiatrie.

déjà une rémunération sur des objectifs de qualité et de permanence des soins, y compris un système de malus

Le présent article tend non seulement à élargir ce dispositif aux hôpitaux psychiatriques d'ici à trois ans, mais également à mettre en place, à partir de 2020, un système de pénalités pour les centres hospitaliers ne parvenant pas à respecter ces critères, tant budgétaires que de qualité. Mes chers collègues, la revendication d'un système de santé plus efficient et plus efficace nous est, à toutes et tous, commune. Mais la méthode punitive du Gouvernement ne saurait être la plus efficace. Si aujourd'hui certains hôpitaux ne peuvent dispenser des soins de qualité, c'est tout simplement parce qu'ils n'en pas les moyens, soit que leurs dotations aient baissé, soit qu'ils aient dû faire des choix de restrictions budgétaires. Ainsi, pénaliser pécuniairement les centres de soins qui ne bénéficient pas des fonds nécessaires à la validation de ces critères de qualité ressemble fortement à

je vous aurais expliqué que la prise en charge du grand âge prend une importance croissante pour tous les acteurs de santé, plus particulièrement pour les 116 800 infirmières libérales, dont 90 % de l'activité est réalisée à domicile et qui visitent quotidiennement 700 000 patients en situation de dépendance, soit 1 % de la population. C'est bien le manque d'organisation autour de la personne âgée, souvent atteinte de polypathologies, et les allers-retours entre l'hôpital et et le domicile qui sont la principale cause de dépenses, conclut dans ses travaux sur le vieillissement le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. Il existe des éléments importants de non-qualité liés au cheminement de ces personnes fragiles : recours inapproprié à l'hôpital, mauvais usage du médicament, manque de réactivité dans l'adaptation des traitements médicamenteux, carences dans l'éducation thérapeutique et la prévention.

En France, l'infirmière de famille apparaît comme le chaînon manquant dans le panorama de la santé publique. Consultation, évaluation de la dépendance, visite de médication, élaboration d'un plan d'aide et de soins, mais aussi coordination sociale et soignante : telles seraient les principales missions de l'infirmière référente.

Il est impératif de proposer des réformes de fond, afin de prendre des mesures financières d'urgence pour certains établissements, de donner un coup d'arrêt dès 2019 à la baisse des tarifs de la régulation prix-volume dans un contexte d'activité stable et de restituer les crédits des établissements de santé non consommés, pour ne plus faire de l'hôpital une variable justement. de prendre des mesures afin de répondre immédiatement à la situation de crise sans précédent, notamment dans la psychiatrie publique, et de réduire les inégalités territoriales en santé. Dans le département des Deux-Sèvres, que je représente, le centre hospitalier de Niort pâtit de ce manque de moyens, notamment dans le service de psychiatrie,

mais avec des problèmes particuliers. Je pense notamment aux personnels de l'établissement du Vinatier, à Bron, qui dénoncent la dégradation des conditions de prise en charge des patients. Je pense également aux personnels du centre hospitalier Alpes-Isère de Saint-Égrève, qui dénoncent la maltraitance institutionnelle,

visent, à chaque fois, à obtenir des postes supplémentaires, tant il est difficile de continuer à prodiguer des soins aux patients avec des moyens restreints.

centré sur le symptôme, en contradiction, selon moi, avec un soin de qualité centré sur le sujet, impliquant une clinique individualisée. C'est vrai en général,

dans les hôpitaux, la qualité de la lettre de liaison à la sortie et la satisfaction des patients hospitalisés. Nous sommes évidemment favorables à la prise en compte de l'avis des patients, qui passe notamment par une démocratie sanitaire revalorisant la place des représentants des usagers au sein des hôpitaux. Mais les critères de validation des indicateurs de qualité et de sécurité des soins sont aujourd'hui détournés pour justifier la fermeture des établissements de santé de proximité. Ces critères ne prennent pas en compte les conséquences des politiques d'austérité en matière de santé menées depuis des décennies et qui ont dégradé

Étendre l'IFAQ aux activités de psychiatrie à partir de 2020 aggravera encore les difficultés rencontrées par les établissements psychiatriques. Alors non, madame la ministre, la transformation du système de soins que vous

qui encourage les établissements à faire mieux dans leurs organisations au bénéfice des patients. L'entrée en vigueur de ce dispositif est fixée au 1 mars 2019. Les indicateurs, qui sont en préparation, seront réévalués tous les trois ans par la Haute Autorité de santé,

intraitable, parce que ce que j'ai vu dans certains hôpitaux est absolument affligeant. Je travaille sur ces trois leviers, mais je ne veux pas que nous nous privions de ces indicateurs de qualité dans nos hôpitaux psychiatriques. Il n'y a aucune raison qu'ils échappent à notre devoir d'améliorer la qualité des soins.

des médecins, des infirmiers et des infirmières. C'est un tout ! On voit là que la psychiatrie est quand même le parent pauvre de la médecine. Il faut une loi

il faut obliger les territoires à avoir un programme de santé mentale coordonné. Nous travaillons aujourd'hui avec les ARS et l'ensemble des professionnels de la psychiatrie, qu'elle soit hospitalière ou libérale,

contre les comportements des personnels préjudiciables aux patientes et aux patients, en particulier dans le domaine gynécologique et obstétrical, ainsi que, d'autre part, la référence au programme relatif à la prévention des violences sexuelles.

consacré un rapport aux actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical, qui a été publié en juin dernier. Notre commission souhaite bien sûr que les recommandations formulées soient mises en oeuvre pour objectiver le phénomène et condamner les pratiques qui doivent l'être, sans jeter néanmoins l'opprobre sur le corps médical dans son ensemble. Le recueil des expériences des patients, qui pourra d'ailleurs y contribuer, de même que les indicateurs transverses de qualité des soins. Toutefois, il n'a pas semblé opportun à la commission de cibler la dotation avec le critère que vous proposez. est donc défavorable. Quel est l'avis du Gouvernement ? Nous sommes évidemment tous concernés par les questions des violences faites aux femmes. Je crois que ce gouvernement a démontré à quel point il était engagé sur la question.

la déclaration sur la satisfaction des patients, c'est-à-dire le dispositif e-Satis, mis en place par la Haute Autorité de santé, lequel est inclus dans les critères de qualité des établissements donnant droit à

Mme Victoire Jasmin. Madame la ministre, mon amendement concerne les démarches de certification et d'accréditation qui sont déjà entreprises par bon nombre d'établissements.

qui sont déjà établis. Malheureusement, ces démarches d'amélioration continue de la qualité sont soumises à des critères qui devraient sans doute être plus pertinents et cohérents

de prévenir et d'intégrer les commissions médicales dans l'élaboration du plan d'amélioration me semble une bonne chose. Je propose donc le retrait de l'amendement de Mme Jasmin au profit de celui de la commission des affaires sociales, auquel je suis favorable.

du Gouvernement ? Madame la sénatrice, je souhaite que mes propos soient bien compris. La situation que vivent nos territoires ultramarins en termes d'accès à la santé est compliquée, particulièrement en Guadeloupe.

est à Mme Laurence Cohen. Dans la suite logique de notre amendement précédent visant à supprimer le dispositif IFAQ, nous proposons de supprimer l'article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale, relatif au contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins, alias CAQES, issu du PLFSS pour 2016. Nous avions déjà, à l'époque, dénoncé cette disposition. En effet, cet article dispose que le contrat a pour objet d'améliorer la qualité, la sécurité et la pertinence des soins et des prescriptions et de permettre une diminution des dépenses de l'assurance maladie. L'objectif, et c'est bien le fil rouge de votre PLFSS,

travailler sur la façon dont nous pouvions évaluer la gestion des ressources humaines et la qualité de vie au travail dans les établissements. Depuis,

présent projet de loi, une double sanction pourrait désormais exister avec le CAQES. J'ai bien entendu vos propos, madame la ministre. Vous nous avez expliqué que les sanctions étaient exceptionnelles et que le risque de double peine était très faible,

ma volonté sera de rendre du temps médical, d'arrêter les usines à gaz et les millefeuilles. Je serai extrêmement attentive à tout ce qui peut recentrer le corps médical sur la pratique de soins. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

chronique. Nous avons commencé par tarifer au forfait le parcours au sein de l'établissement, parce que nous étions prêts. Nous avions délimité ce que devait être le parcours de soins dans l'établissement.

durée. L'intention développée à l'article 28 de garantir une meilleure prise en charge des pathologies chroniques, par-delà l'épisode aigu, en prévention de son apparition, constitue un progrès significatif. L'incitation des professionnels et des structures à développer les actions de prévention, d'éducation du patient et à assurer et à assurer la fonction de coordination des soins est aujourd'hui indispensable pour assurer une prise en charge de qualité et un parcours de soins plus efficient. Les patients atteints de pathologies chroniques reconnues par la sécurité sociale comme affection de longue durée, ou ALD, et requérant le diagnostic et le suivi de multiples spécialistes pourraient grandement bénéficier de cette initiative.

projet de loi comprend un certain nombre de mesures destinées à transformer la prise en charge des patients souffrant de maladies chroniques, et notamment, donc, d'insuffisance rénale chronique.

plus efficientes » et notait que « les modalités qui favorisent une meilleure qualité de vie ne sont pas assez développées » et que leur développement pourrait dégager des marges de manoeuvre financières importantes pour la sécurité sociale. Dans ce contexte, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, 2019, comme le plan « Ma santé 2022 », ouvre de nouvelles perspectives : il prévoit dès 2019 la création de financements au forfait pour la prise en charge à l'hôpital des pathologies chroniques, dont l'insuffisance rénale. L'article L. 162-22-6-2 inséré dans le code de la sécurité sociale prévoit une rémunération forfaitaire des prestations, dans le cadre d'un parcours de soins, pour la prise en charge des patients atteints d'une pathologie chronique. Dès 2019, la prise en charge de l'insuffisance rénale sera assurée par ce nouveau mode de financement. Toutefois, ce nouveau dispositif incitera les établissements de santé à privilégier les prises en charge les plus lourdes, qui sont aussi les plus rémunératrices. Par conséquent, afin d'éviter une telle situation, à la fois pour le confort des patients et

Il existe aujourd'hui plusieurs parcours de soins possibles et les circonstances font que, en France beaucoup plus que dans les autres pays, c'est le parcours de soins le plus coûteux, le plus lourd, et celui qui, en définitive, a le plus de conséquences sur la vie des patients, qui est retenu. Il est donc nécessaire que nous puissions prendre des dispositions

je regrette, madame la ministre, que le Gouvernement n'aille pas au bout de sa logique en appliquant dès 2019 la forfaitisation à l'ensemble des parcours, y compris, donc, à la transplantation et à la dialyse. En effet, 85 % des dépenses liées à cette pathologie, ce qui représente quand même près de 4 milliards d'euros pour l'assurance maladie, concernent la dialyse et les transports transports liés aux traitements les plus lourds- je rejoins, de ce point de vue, Yves Daudigny. Le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, dans son rapport de 2016, note que « les établissements souhaitent avant tout " remplir " leur centre de dialyse ». Les tarifs sont en effet très favorables au développement des thérapies les plus lourdes et les plus coûteuses. Une baisse uniforme des tarifs de dialyse conduirait à accentuer ce biais. La Cour des comptes, dans son rapport sur l'insuffisance rénale chronique terminale de septembre 2015, préconise le développement de la greffe et de la dialyse à domicile. est aussi la conclusion de l'évaluation médico-économique des stratégies de prise en charge de l'insuffisance rénale chronique terminale en France réalisée par la Haute Autorité de santé en 2014. Il est donc essentiel, madame la ministre, que la baisse annoncée des tarifs de dialyse épargne la dialyse à domicile, afin de maintenir cette option thérapeutique qui correspond à l'intérêt des patients et à celui de l'assurance maladie.

quand pensez-vous ouvrir la forfaitisation à la dialyse et à la greffe ? La parole est à Mme la ministre.

je souhaitais attirer votre attention sur un problème de santé très présent dans le territoire dont je suis l'élu, Paris, à savoir l'épidémie d'infections sexuellement transmissibles, et notamment la permanence de l'épidémie de VIH. Nous avons organisé, ici, au Sénat, au mois de juin, des rencontres nationales avec les différents acteurs des territoires les plus concernés, l'Île-de-France, les territoires ultramarins, la région PACA, sur les outils à mettre en oeuvre pour mettre fin à l'épidémie de VIH, qui stagne depuis un certain nombre d'années.

et le dépistage : ce délai est en moyenne de quatre ans pour les hommes hétérosexuels, de trois ans pour les femmes et de deux ans pour les hommes ayant des rapports avec d'autres hommes.

on sait ce qui se fait à Londres ou aux États-Unis -afin de simplifier l'accès au dépistage et à une prise en charge globale des infections sexuellement transmissibles. Je souhaitais attirer votre attention,

sans grand succès jusqu'à présent. Je pense notamment au système de coopération entre les professionnels de santé testé par plusieurs agences régionales de santé, qui peine à trouver son chemin- et c'est bien fait. La solution

Il va de soi qu'il n'est pas question de laisser les optométristes accomplir quelque travail thérapeutique ou de diagnostic que ce soit.

Ce dispositif d'innovation avait pour objectif de permettre l'émergence d'organisations innovantes dans les secteurs sanitaire et médico-social et de favoriser une prise en charge pertinente de la part de l'assurance maladie. L'objectif était, entre autres, d'améliorer l'accès aux soins dans les zones médicalement sous-dotées. Vous vous en doutez : nous soutenons ce dernier nous nous sommes opposés, il y a un an, à ce cadre d'expérimentation, et nous nous opposons à son extension cette année. En effet, le cadre d'expérimentation adopté l'an dernier prévoyait la suppression de l'opposabilité des conventions collectives de travail dans les établissements et services du social et du médico-social, ainsi que la possibilité de déroger aux règles de rémunération et d'organisation des services. Cet article 29 confirme cette volonté de dérégulation ; il prévoit la possibilité de déroger aux conditions techniques de fonctionnement, c'est-à-dire aux normes applicables aux organisations, aux équipements, aux locaux, aux ratios de personnel. Nous considérons que l'amélioration de la prise en charge des plus fragiles et la lutte contre les déserts médicaux ne doivent pas se faire au détriment des personnels de santé. La lutte contre les déserts médicaux passe, d'une part, par l'augmentation des financements permettant la création de centres de santé et l'embauche de personnels, et, d'autre part, par des dispositifs incitant les médecins à s'installer dans les zones sous-dotées. Par « incitation », nous ne parlons pas de permettre aux médecins salariés de travailler en libéral, comme cela est proposé dans cet article. Cette mesure injuste permet aux médecins de cumuler deux rémunérations sans pour autant installer de médecine de proximité stable. Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article. Quel

Mme Préville, est ainsi libellé : La parole est à Mme Angèle Préville. À l'alinéa 4, le Gouvernement propose d'étendre les possibilités d'exercice libéral pour les praticiens hospitaliers salariés d'un hôpital public, dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante. insuffisante. L'article ne précise pas comment ces zones sont caractérisées, ce qui laisse un flou législatif qui peut conduire à des excès. En outre, un problème non négligeable demeure : les données publiées

Afin d'analyser la part d'activité libérale par rapport à l'activité publique, il est nécessaire que les données d'activité publique soient connues. La CCAL note encore à de trop nombreuses reprises la difficulté rencontrée [ ...] à répertorier l'activité publique. La CCAL souhaite que ces difficultés soient rapidement levées et être informée des dispositions prises pour assurer un suivi de l'activité publique des praticiens exerçant une activité libérale. » Ce commentaire illustre les difficultés de suivi du respect des obligations prévues par la loi, s'agissant en particulier du non-dépassement d'honoraires,

celle-ci. Cet amendement a donc pour objet de préciser le dispositif. Nous croyons qu'il y a là une piste immédiatement applicable, en attendant les effets du plan « Ma santé 2022 », dont il rejoint la philosophie, avec la mise en place d'assistants médicaux. permettrait d'expérimenter un exercice libéral simplifié à partir d'un centre de santé. Les jeunes médecins y trouveraient d'importants facteurs d'attractivité : il s'agit d'un mode d'exercice médical en équipe, qui ne nécessite pas d'installation ni n'impose de contraintes immobilières, informatiques, administratives ou de gestion des personnels affectés. Cette expérimentation permettrait aussi de gagner du temps médical avec le patient, de l'ordre de 40 % par médecin, améliorant d'autant l'accès aux soins pour les très nombreux patients n'ayant aujourd'hui pas de médecin traitant.

derniers a acté qu'ils étaient exclusivement en exercice salarié. Aujourd'hui, rien n'empêche un professionnel libéral d'exercer à mi-temps sous la forme d'exercice salarié dans un centre de santé et à mi-temps en libéral à l'extérieur, voire dans une maison de santé pluriprofessionnelle. Nous ne souhaitons pas

adapter la posologie, en concertation étroite avec le médecin traitant. Cette expérimentation peut être fort utile dans les territoires touchés par la désertification médicale. L'infirmier, qui intervient le plus souvent à domicile, est tout à fait qualifié pour exercer un tel suivi quotidien, surveiller l'observance du traitement et recueillir des informations cliniques utiles. Afin de garantir une bonne collaboration avec le médecin prescripteur, ces infirmiers devront être adhérents ou signataires du projet de santé d'une maison de santé pluriprofessionnelle ou d'une équipe de soins primaire. La parole est à M.

Le nouveau champ d'expérimentation ouvert sur l'initiative de l'Assemblée nationale reprend une possibilité qui existe déjà pour les pharmaciens d'officine. Un protocole de coopération avait été

du Gouvernement ? Les infirmières de pratique avancée qui se sont inscrites en master à partir de 2019 auront la possibilité, dans leurs missions, d'effectuer des renouvellements d'ordonnance. Cela fait aujourd'hui partie du champ d'investigation des pratiques avancées dans le cadre de coopérations avec les médecins.

place des infirmières est entière dans la réforme « Ma santé 2022 », notamment pour le suivi des pathologies chroniques. Mais, pour l'instant, nous n'avons pas franchi le cap des prescriptions. Nous préférons attendre de voir ce que donneront les pratiques avancées. Le Gouvernement

a pour objet d'établir un cadre temporel raisonnable pour le renouvellement des traitements chroniques par les pharmaciens. Seul le médecin traitant doit pouvoir ajuster la posologie des traitements des patients atteints de pathologies chroniques. Quel est l'avis de la commission

organisationnelles et de permettre d'expérimenter de nouvelles formes de coopération entre les acteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires au service du parcours de santé et de vie des personnes d'autre part, les modalités de qualification entre actes d'aide et actes de soins dans le cadre d'un accompagnement par un établissement ou service social ou médico-social. Sur ce deuxième point, l'actuel cloisonnement des métiers de l'aide et du soin conduit à une étanchéité des missions, en particulier à domicile, entre aide à domicile, titulaire du d'accompagnant éducatif et social, et aide-soignant, titulaire du diplôme d'État d'aide-soignant. Ce cloisonnement obère la qualité et la pertinence de l'accompagnement dans son objectif de préservation ou de renforcement de l'autonomie des personnes dépendantes d'un tiers pour la réalisation de gestes de soins rendus nécessaires du fait d'un handicap ou de l'avancée en âge. Par ailleurs, les acteurs développent aujourd'hui des organisations complexes et coûteuses en coordination pour compenser ce cloisonnement des métiers de l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie. de nouvelles répartitions entre actes d'aide et actes de soins en fonction des besoins des personnes elles-mêmes, lors d'un accompagnement par un établissement ou service social ou médico-social, il sera possible d'identifier les « fongibilités de compétences » sociales et de soins en fonction des situations. La parole

Mais nous prenons en compte le fait que l'article 29 ajoute déjà aux règles de tarification celle d'organisation dans les possibilités de dérogation à l'alinéa 9, afin de pouvoir ainsi développer des expérimentations organisationnelles dans le secteur médico-social. vise ainsi à étendre les possibilités de dérogation prévues à l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale pour l'expérimentation dans le secteur sanitaire et médico-social et à permettre des délégations de soins en matière d'aide et d'éducation des personnes porteuses de handicap et également de soins infirmiers. Cela permettra notamment de dépasser les cloisonnements entre aide et soins dans l'accompagnement à l'autonomie des personnes dépendantes du fait d'un handicap ou de l'âge.

Cela touche directement la définition des métiers d'aide-soignant et d'aide à domicile. Pour nous, une telle mesure se prête mal à une expérimentation locale et nécessite une réflexion plus globale que nous aurons sur ces professions dans le cadre de la de la consultation sur les métiers de la perte d'autonomie. Nous travaillons aux évolutions potentielles des métiers et à d'éventuelles délégations de tâches. Je ne souhaiterais pas accompagner des expérimentations dans ce champ. Je sollicite donc le retrait de

à l'augmentation importante des maladies chroniques. C'est également un enjeu financier, comme l'ont montré les travaux sur le vieillissement du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. maladie. Les recours inappropriés à l'hôpital, le manque de réactivité dans l'adaptation des traitements médicamenteux ou le manque de prévention et d'éducation thérapeutique appellent de nouvelles réponses. Nous avons du mal à opérer la mue de notre système de soins pour accompagner qualitativement le cheminement des personnes fragiles. Alors que, en France, nous cherchons à inventer de nouveaux métiers autour du soin, nous voyons que les infirmières demeurent un chaînon insuffisamment reconnu du panorama

Il permet de redonner au chaînon que sont ces professionnels toute leur importance pour la qualité et l'efficacité dans la prise en charge des personnes. Je crois que cette mesure marquerait un pas non négligeable dans l'évolution stratégique de notre système de soins vers davantage de coordination, de reconnaissance des complémentarités au sein des équipes de soins, de qualité et d'efficacité dans le suivi des personnes. Quel

Aujourd'hui, la prévention des hospitalisations et la prise en charge des parcours complexes coordonnés reviennent- c'est le changement de paradigme que nous souhaitons opérer avec la transformation du système de santé -à charger des communautés de professionnels

de soins infirmiers. Il s'agit d'améliorer l'évaluation par l'infirmier des besoins en soins de patients dépendants. Nous pensons que c'est la voie du dialogue entre l'assurance maladie et les syndicats de représentants des infirmiers qui sera privilégiée pour envisager le devenir de cette expérimentation. L'une des missions des communautés professionnelles de territoires de santé que nous créons est le maintien à domicile des personnes âgées polypathologiques. Pour nous, dans ces communautés professionnelles territoriales de santé, les infirmiers libéraux auront leur rôle à jouer autour de cette mission spécifique et de l'organisation dédiée. Nous venons de créer les infirmiers de pratique avancée, qui répondent en partie à une telle préoccupation. Leurs compétences sont élargies et ils auront la responsabilité du suivi régulier des pathologies chroniques. Il nous apparaît donc préférable d'évaluer le bilan de soins infirmiers, c'est-à-dire l'expérimentation, de soutenir de façon volontariste le déploiement des infirmiers de pratique avancée et de renforcer tous les dispositifs de coordination déjà existants, au lieu de créer un nouveau statut, ne correspond pas à notre philosophie. Nous pensons que les infirmiers, notamment les infirmiers libéraux, sont indispensables à la transformation. Ils auront toute leur place dans le dispositif de soins coordonnés, mais nous ne l'envisageons pas sous l'angle de l'infirmier référent.

avec le médecin traitant et le pharmacien correspondant. Vous avez accepté à l'Assemblée nationale cette expérimentation sur le pharmacien correspondant. Il s'agit non créer un nouveau statut, mais de prendre acte du fait que le pharmacien est de plus en plus- c'est heureux -un acteur de santé essentiel dans la coordination du parcours autour du patient. Il est légitime de reconnaître,

une référence unique. Mais nous voulons envoyer le message que c'est bien dans l'articulation de ces trois professions de santé de proximité que se joue

L'intégration dans le droit commun tarifaire des actes de télémédecine et de téléconsultation est une excellente option. Pour autant, il est indispensable que cette thématique nouvelle, créatrice de liens renouvelés entre la ville et l'hôpital, au service des parcours de soins et de vie des patients à domicile, associe d'emblée les professionnels libéraux et hospitaliers et les fédérations hospitalières représentatives, publiques et privées.

négocié cette année entre l'UNCAM et les représentants des médecins pour inscrire les actes de télémédecine dans le droit commun. Il ne semble pas dès lors opportun d'instituer, alors que ces négociations sont passées, une telle commission nous avions jugé l'an passé que ce fonctionnement, calqué sur celui des équipements matériels lourds, était sans doute trop contraignant. S'il importe de ne pas laisser de côté l'hôpital dans la mise en oeuvre de la télémédecine, l'instauration d'une telle commission ne paraît pas, toutefois, le moyen le plus approprié. La commission demande donc le retrait de cet amendement. À

à assurer une composition paritaire des commissions de contrôle de la tarification à l'activité, entre représentants des financeurs et des fédérations hospitalières publiques et privées, à l'instar du dispositif existant pour les professionnels de santé libéraux, afin de favoriser la compréhension et la diffusion optimale de l'information entre les parties prenantes, tout en garantissant tant la justesse que la légitimité des avis produits. Le dispositif de contrôle de la tarification à l'activité est marqué d'imperfections significatives et de déséquilibres sérieux. Cette situation nourrit de très nombreux contentieux et alimente en permanence des discussions intenses entre les fédérations hospitalières publiques et privées, d'une part, et les pouvoirs publics, d'autre part. Le présent amendement a pour objet d'apporter une contribution apaisante au débat, en prévoyant que la commission de contrôle compétente pour avis soit constituée à parité de représentants des financeurs

La commission de contrôle de la T2A, composée de représentants de l'ARS et de l'assurance maladie, est saisie pour avis par l'ARS avant de prononcer toute sanction en cas de manquement aux règles de facturation ou d'erreur de codage.

Les fédérations hospitalières sont associées au processus de contrôle dans d'autres cadres, parce qu'elles sont membres de l'Observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée, qui examine l'application du contrôle de la T2A et les problématiques qu'il soulève sur un plan générique non au moment de chaque contrôle. Elles sont également associées à la révision du guide de contrôle externe de la T2A et elles sont surtout invitées à participer à une réunion de présentation du plan de contrôle en amont du lancement des campagnes de contrôle. En tout état de cause,

après l'article 29. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune. L'amendement n° 394 rectifié,

Laisser les frais et la gestion des transports entre les établissements à la charge des hôpitaux et des autres établissements de santé engendre de grandes difficultés. En outre, un tel dispositif a un impact financier négatif et s'accompagne d'une importante perte de temps. Par conséquent, il doit être supprimé. Les trois

L'article 80 de la loi du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 a introduit l'article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale aux termes duquel tous les transports inter-établissements devraient être pris en charge par les établissements de santé, en lieu et place d'une facturation directe à l'assurance maladie. Force est de constater que cette réforme radicale n'a pas suffisamment été anticipée. Ce désengagement de la solidarité nationale crée des inégalités importantes en fonction des territoires et des établissements concernés. Le coût ne sera pas le même en ville qu'à la campagne. Certains établissements font directement payer les transports aux familles. Or ces dernières ne disposent pas toujours des moyens suffisants. Cet amendement vise à prévoir que ce montant figure expressément dans les arrêtés relatifs aux dotations et tarifs

principe selon lequel tous les transports inter-établissements devraient être pris en charge par les établissements de santé. Cette réforme radicale du financement des transports inter-établissements, entrée en vigueur le 1 octobre 2018, n'a pas été suffisamment anticipée en amont et crée des inégalités importantes entre les établissements concernés. concernés. Cet amendement tend à prévoir, d'une part, que ce montant figure expressément dans les arrêtés relatifs aux dotations et tarifs de tous les établissements de santé et, d'autre part, qu'une évaluation du dispositif permette de revoir les tarifs calculés en 2018.

L'enjeu mis en avant est de mieux structurer la commande et de favoriser une meilleure adéquation entre le type de transport et l'état de santé. Nous ne pouvons qu'y adhérer. Pour la sécurité sociale, indéniablement, c'est une source d'économie qui sera toutefois transférée sur les établissements.

craignent en effet que le compte n'y soit pas. La situation particulière des hôpitaux de proximité, éloignés des centres techniques, doit être prise en compte. la crainte des entreprises de transport, notamment les plus petites d'entre elles, qui seront soumises à des appels d'offres sur un segment de leur activité. Elles devront ainsi face aux grosses

précise de son impact financier seraient en effet souhaitables. Nous attendons parallèlement de votre part, madame la ministre, des précisions sur les modalités de ce transfert et sur son suivi, notamment en ce qui concerne l'accompagnement proposé aux établissements de santé.

? Je rappelle qu'il n'y a aucun désengagement en termes de solidarité nationale sur la question du transport sanitaire. Il y a juste eu transfert d'une enveloppe budgétaire de la CNAM vers les établissements

réforme fait l'objet d'un suivi, d'une part, avec les fédérations hospitalières et, d'autre part, avec les fédérations de transporteurs. Nous avons prévu un comité de suivi

à l'ensemble de ces amendements. C'est une réforme qui se met en oeuvre, elle est très importante pour les établissements de santé et la rationalisation des transports entre établissements.

: La parole est à Mme Monique Lubin. Le comité technique de l'innovation en santé est composé de huit membres représentant la Caisse nationale de l'assurance maladie, le secrétariat général des ministères sociaux, les directions du ministère chargé de la santé et des agences régionales de santé. Il émet un avis sur les projets d'expérimentation qui lui sont soumis, sur leur mode de financement, ainsi que sur leurs modalités d'évaluation. Ce comité doit également saisir pour avis la Haute Autorité de santé lorsque les projets d'expérimentation comportent des dérogations à des dispositions du code de la santé publique relatives à l'organisation ou à la dispensation des soins. Il est en outre destinataire des rapports d'étape rédigés par les porteurs de projet et des rapports d'évaluation sur la base desquels il rend un avis sur l'opportunité et les modalités d'une généralisation. Le présent amendement vise à assurer une représentation plus juste et plus équilibrée au sein du comité technique de l'innovation en santé afin que les différents cofinanceurs de l'action médico-sociale puissent y figurer et participer à ses travaux. C'est la raison pour laquelle il est proposé d'associer aux travaux du comité technique de l'innovation en santé des acteurs de l'assurance vieillesse, des représentants des conseils départementaux et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, ainsi que la conférence des financeurs mentionnée à l'article L. 233-1 du code de l'action sociale et des familles, compétente en fonction de la territorialité du projet. De la sorte, dans un esprit respectueux du principe de décentralisation et des spécificités de chaque secteur d'intervention concerné, il sera possible de promouvoir des expérimentations répondant effectivement à des besoins identifiés, selon des modalités qui en garantissent les meilleures chances de succès pour un coût adapté. pour un coût adapté. Quel est l'avis de la commission ? Nous avions eu ce débat l'an passé, et nous avons considéré que le comité technique de pilotage des expérimentations devait rester restreint, tandis que le conseil stratégique avait un champ plus large installé en début d'année, ce conseil stratégique compte un représentant de la CNSA, un autre de l'ADF et des acteurs du champ médico-social. Au niveau régional, la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie placée auprès des ARS doit être consultée, comme nos débats l'avaient mis en évidence.

Cet amendement vise à offrir la possibilité aux fédérations hospitalières de devenir porteuses de projets d'expérimentation dont les modalités sont renvoyées à un arrêté ministériel, de sorte que le Gouvernement puisse établir un mécanisme conforme aux aspirations de la réforme. Ainsi, l'innovation dans le système de santé sera davantage motivée. La parole

162-50-5 et suivants du code de la sécurité sociale puissent répondre et candidater à un projet d'expérimentation. Cela favoriserait le succès du dispositif comme son appréhension par les acteurs du système de santé.

par un professionnel de terrain. Les fédérations sont largement représentées dans tous les projets, elles les cogèrent avec les professionnels, mais nous ne souhaitons pas un portage

à Mme Corinne Imbert. La présente proposition de modification législative vise à soumettre pour avis préalable aux fédérations hospitalières publiques et privées les mesures conventionnelles qui ont des répercussions significatives sur le pilotage et la gestion des établissements de santé, dans le cadre des concertations précédant le précédant le mécanisme d'approbation tacite ou d'opposition expresse du ministre chargé de la sécurité sociale. La loi du 13 août 2004 confie aux représentants des médecins libéraux et à l'UNCAM le soin de hiérarchiser et de fixer les tarifs des actes médicaux. Les fédérations hospitalières ne sont pas consultées ni même parfois informées des discussions engagées dans ce cadre alors qu'elles sont directement concernées par les résultats de ces négociations. En effet, elles ont un impact dans la construction du PMSI et sa valorisation dans le cadre de la tarification à l'activité, qui repose sur la classification commune des actes médicaux. En outre, la valorisation des actes médicaux a des conséquences directes sur les choix d'exercice des médecins entre une pratique dans le secteur libéral et une pratique à l'hôpital public. Cela est d'autant plus vrai que la loi permet aux médecins libéraux d'être employés dans les établissements publics de santé. Dans ce contexte, il importe que les fédérations hospitalières puissent être concertées en amont de l'élaboration des conventions annexes et des avenants conclus entre l'UNCAM et les professionnels de santé.

et les professionnels de santé qui vont négocier au sein de la convention avec la CNAM.

santé. Je comprends la nécessité pour les gestionnaires d'établissements d'anticiper les conséquences des accords conventionnels passés avec les professions libérales, par exemple sur les actes et les tarifs des consultations externes. Toutefois, ces modalités de transposition des évolutions de tarifs des actes pour les établissements de santé sont d'ores et déjà clairement définies par les textes réglementaires. En outre, les négociations conventionnelles ne sont rendues publiques et n'entrent en vigueur que six mois après la signature de l'accord, ce qui permet d'anticiper toute évolution.

En effet, l'absence de publication de l'arrêté tarifaire à cette date règlementaire empêche les caisses primaires d'assurance maladie d'accepter les factures émises pour les patients à compter du 1 mars de l'année concernée, tant que la nouvelle classification n'est pas publiée. Selon les années, des dispositifs d'avances sont consentis sur l'initiative des caisses ou à la demande des établissements. Cependant, en l'absence d'une disposition législative pérenne et claire, cette situation met chaque année

embellie. Quel est l'avis de la commission ? Ces amendements visent à remédier aux difficultés financières rencontrées par des établissements de santé du fait de la publication avec retard de l'arrêté tarifaire, en uniformisant des pratiques.

concernant un GHT la veille de la prise de fonctions du directeur de l'ARS dans une autre région. Cet amendement a pour objet de renforcer la coproduction en amont,

en réalité, cela existe déjà, et je vais vous expliquer comment nous procédons. Aujourd'hui, les ARS produisent un rapport annuel du FIR,

En parallèle existent des indicateurs de santé par région qui sont publiés par Santé publique France. Nous croisons toutes ces données lorsque nous établissons un projet régional de santé. Je vous rappelle que le PRS est négocié avec l'ensemble des parties prenantes, sur la base

Une tendance au renforcement des missions de prévention et de coordination des parcours est d'ailleurs observée, elle est lisible. Par ailleurs, chaque ARS produit annuellement un rapport d'activité qui comporte les éléments relatifs à la gestion des crédits alloués dans le cadre du Fonds d'intervention régional.

du code de la santé publique, les structures autorisées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation complète « sont tenues d'organiser la continuité des soins en dehors de leurs heures d'ouverture, y compris les dimanches et jours fériés Les structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit et les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires doivent ainsi s'organiser en interne pour ce faire. pour ce faire. Dans le cas où l'une de ces structures ne serait pas en mesure d'assurer elle-même la continuité des soins, le même article prévoit qu'« elle qu'« elle est tenue de conclure une convention avec un autre établissement de santé accueillant en hospitalisation à temps complet des patients relevant de la ou des disciplines pratiquées par la structure Cette disposition limite inutilement aux seuls établissements autorisés en hospitalisation complètela participation à la continuité des soins des patients admis dans des structures alternatives à cette même hospitalisation complète. Le présent amendement vise donc à favoriser leur implication dans cette prise en charge, afin qu'ils puissent contribuer, au même titre que les autres établissements de santé, à la continuité des soins des patients admis initialement dans les structures autorisées.

suffisamment sécurisé pour le patient, afin qu'il ne soit pas nécessaire d'assurer un relais une nouvelle hospitalisation, y compris en HAD. Ce que vous proposez est donc quelque peu antinomique

C'est un outil indispensable pour caractériser la politique de santé mise en oeuvre par les gouvernements successifs. Ce document met en évidence leurs priorités et permet de se confronter aux conséquences des grandes orientations adoptées. Il s'agit aussi d'une incitation à faire évoluer ces politiques et à les réviser si besoin est. Les éléments qui sont présentés ne sont cependant plus suffisants pour avoir une bonne appréciation de l'évolution de la situation des personnels. On observe en effet qu'une inquiétude grandit sur leurs conditions de travail, lesquelles ne peuvent qu'impacter la qualité de l'offre de soins et d'accompagnement. Le manque de moyens humains dont souffrent les établissements de santé fragilise ainsi la confiance des patients en un système de santé et un monde hospitalier qui demeurent pourtant remarquablement performants, et ce malgré l'extraordinaire pression à laquelle ils sont soumis. Les conditions dégradées dans lesquelles travaillent les personnels, trop souvent débordés, en sous-effectif, confronté au et, plus généralement, victimes d'une fatigue morale et psychique, ne peuvent qu'altérer, à terme, leur capacité à mener leurs missions, malgré tout le dévouement du monde. C'est la raison pour laquelle les acteurs du secteur réclament une évolution des politiques de ressources humaines en direction de ces personnels de santé qui soit orientée dans le sens d'une véritable politique sociale. Il s'agit aussi de promouvoir des parcours professionnels cohérents, construits, qui fassent sens, permettent l'épanouissement des personnels et favorisent l'accomplissement de leur mission dans les meilleures conditions possible. Pour ce faire, il est indispensable de disposer d'une photographie la plus précise possible des conditions dans lesquelles s'effectue leur parcours professionnel. Dans cette optique et dans l'objectif d'améliorer l'information et le contrôle du Parlement sur l'évolution des dépenses de personnels des établissements de santé, nous proposons d'annexer à la loi de financement de la sécurité sociale le chiffrage des mesures catégorielles relatives aux personnels médical et non médical. Les acteurs professionnels concernés doivent aussi pouvoir bénéficier de cette amélioration de l'information en ayant accès à ce chiffrage lors de la consultation des instances nationales de dialogue social.

L'article 29 , issu d'un amendement du Gouvernement, affiche l'objectif louable de « dynamiser » les actions conduites dans le domaine de la pertinence des soins. Ce faisant, il introduit un nouvel instrument, le programme d'amélioration de la pertinence des soins, dont on comprend mal l'articulation avec les outils existant déjà pour intervenir auprès des établissements identifiés pour leurs pratiques « atypiques à savoir notamment la conclusion d'un volet additionnel au CAQES, le contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins. L'amendement vise donc à clarifier l'articulation entre ces outils.

L'amendement que vous proposez vise à préciser que le nouveau programme d'amélioration de la pertinence des soins sert de base à la mise en place d'un volet additionnel. Dans les faits, les données qui servent à l'établissement du programme d'action et à un éventuel CAQES sont les mêmes, et les deux procédures sont complémentaires. L'amendement viserait donc à systématiser

de cause. Les établissements concernés devraient pouvoir patienter encore quelques semaines avant de restructurer leur dette, leur cas n'ayant, par définition, pas été traité depuis le lancement du premier plan d'aide, en 2014.

Je vous rappelle qu'une mesure identique avait été prévue pour les collectivités locales dans le cadre de la loi de finances et qu'elle n'avait pas été censurée par le Conseil constitutionnel. Sur le fond, le Gouvernement tient beaucoup à cette disposition importante pour les hôpitaux qui connaissent une situation financière très difficile. Près d'une centaine d'hôpitaux sont concernés, pour un montant représentant environ 450 millions d'euros de dettes toxiques, c'est-à-dire plusieurs millions d'euros

à risque et dans quelles conditions, quels établissements seraient concernés par le nouveau dispositif, pour quel montant de prêt et pour quel niveau maximum de taux, et si les établissements pourront bénéficier de l'expertise de la Banque de France pour sécuriser leur emprunt emprunt dans les meilleures conditions financières. Nous n'avons pas non plus de comparatif de la situation financière qui résulterait, pour un établissement type donné, de la conversion des indemnités de remboursement anticipé en montant d'un nouvel emprunt

Oui, cela nous concerne

Il me semble donc anormal que, pour les hôpitaux, ce soit à l'assurance maladie de prendre en charge les investissements immobiliers. Il serait plus logique que ce soit

aucune discussion n'a eu lieu afin de s'interroger sur l'opportunité d'une telle création ou sur son articulation avec les professions existantes. Cet amendement vise donc à supprimer le présent article dans l'attente d'études plus approfondies.

Ainsi, la création récente des assistants dentaires a été introduite par la loi de 2016 de modernisation de notre système de santé, qui a fixé le cadre de compétences et prévu les dérogations à l'exercice illégal de l'art dentaire. Or, dans le cas présent, l'article 29 se contente de renvoyer à une convention entre l'assurance maladie et les médecins le soin de définir le cadre de compétences de cette profession. Cette disposition escamote toute concertation avec le Parlement, ainsi que toute concertation avec les autres professions de santé qui peuvent pourtant être sérieusement affectées par la création de ce nouveau métier.

L'année dernière, madame la ministre, vous m'aviez répondu qu'il était difficile de dresser une carte précise des secteurs sous-dotés, surdotés ou normalement dotés.

Dans le contexte de désertification médicale que connaît notre pays, la création de cette profession ne me semble pas de nature à constituer une solution. Une extension du champ des pratiques avancées, définies dans un décret récent au profit des professionnels de santé déjà habilités, constituerait bien davantage un progrès en déchargeant les médecins d'actes qu'ils n'ont pas toujours le temps de réaliser. ministre, le mécontentement des territoires ne porte pas uniquement sur la fiscalité, mais sur la première préoccupation des Français : l'accès aux soins. On ne peut plus accepter la situation actuelle, qui ne fait que se dégrader. Au Sénat, nous sommes attachés aux territoires et devons collectivement être courageux dans nos propositions. Je le dis notamment à mes collègues qui sont sénateurs et médecins.

mission auprès d'eux, de façon à pouvoir recentrer le temps médical sur ce qui a une forte valeur ajoutée. Aujourd'hui, nous avons un déficit de temps médical sur tout le territoire. Le nombre de postes créés correspond en gros à 4 000 postes dédiés à des exercices

Quels sont les professionnels qui pourront s'inscrire ? L'idée n'est évidemment pas de faire concurrence à des professions de santé existantes. Les infirmières ont des rôles évidemment bien supérieurs, bien plus larges que ce que pourrait être la mission des assistants

Aujourd'hui, il existe des zones sous-dotées identifiées par zonage, qui figurent évidemment dans la cartographie des régions et permettent d'être incitatives. Toutefois, nous pensons que ces professionnels auront vocation à se rendre partout sur le territoire pour des exercices regroupés.

nous vous faisons confiance pour cette nouvelle mission. C'est l'esprit qui a animé la commission, et nous aurons, je pense, l'occasion d'en reparler. C'est pourquoi je ne voterai pas les amendements de suppression.

Vous prévoyez toutefois dans la loi une condition impérative, à savoir l'exercice coordonné. Quand le chef de l'État a rendu public sa décision de créer des assistants médicaux

coopération avec les autres professionnels », sans s'inscrire dans une démarche de parcours de soins coordonné ne peut plus être l'avenir de la médecine.

de participer à des délégations de tâches, de mieux travailler avec les infirmières, les kinés, les pharmaciens puissent bénéficier plus facilement d'aides que ceux qui restent dans un exercice

Il ne serait pas acceptable que, tel que le laisse pressentir la rédaction actuelle de l'article, avec les termes « modulation » et « cadre d'exercice », seules certaines formes d'exercice coordonné se voient valorisées. Le nouvel accord-cadre interprofessionnel, signé le 10 octobre 2018 entre l'Union nationale des professionnels de santé et l'assurance maladie, prévoit, outre la mise en oeuvre des dispositifs issus de la loi du 26 de santé, le développement d'autres formes d'organisations pluriprofessionnelles capables d'apporter une réponse coordonnée de proximité aux besoins de prise en charge des patients. Je citerai, notamment, les équipes ouvertes non formalisées de professionnels de santé libéraux. Ainsi, tout professionnel de santé engagé dans une prise en charge coordonnée, quel que soit son mode d'exercice, doit recevoir une rémunération en sus pour le temps dédié à cette coordination. Le présent amendement tend donc à ouvrir la rémunération de la coordination à l'ensemble des professionnels de santé.

leurs conventions avec l'assurance maladie, à développer les prises en charge coordonnées. Or, tel qu'il est rédigé, seules certaines formes d'exercice coordonné seraient valorisées. Aussi, par cet amendement, qui rejoint celui de Mme Micouleau, nous proposons d'ouvrir la rémunération de la coordination à l'ensemble des professionnels de santé. Nous estimons en effet que tout professionnel de santé engagé dans une prise en charge coordonnée, quel que soit son mode d'exercice, doit recevoir une rémunération en sus

l'esprit dans lequel nous construisons le système de santé de demain. Nous souhaitons que les professionnels s'inscrivent dans un cadre donné, notamment les CPTS, qui

citoyen un médecin traitant, de proposer une permanence des soins non programmés et

et à l'échelle des bassins de vie. Je suis opposée à ce changement sémantique, car, derrière, c'est un véritable changement structurel que vous feriez vivre à la réforme que je souhaite mener.